La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 30 octobre 2024 a été publié sur le site internet du Sénat.

Plusieurs entreprises, autrefois piliers de l’emploi local, sont aujourd’hui en proie à de graves difficultés financières. Je dois évidemment évoquer la situation de la papeterie Stenpa, à Stenay, où 130 emplois sont menacés. Moins d’un an après sa reprise par un fonds d’investissement étranger, cette papeterie quasi centenaire se retrouve une nouvelle fois au bord du gouffre, puisque les promesses d’investissement n’ont pas été tenues. À cela s’ajoute un nouveau coup dur pour l’emploi local et le tissu économique meusien avec l’annonce de la fermeture par Bonduelle de son site de Saint Mihiel, où 159 salariés risquent de perdre leur travail. Sans un engagement fort de l’État pour identifier et accompagner des repreneurs, la désindustrialisation des territoires ruraux ne pourra être stoppée. Dans des territoires comme la Meuse, où l’industrie constitue le dernier rempart contre l’exode rural, ces fermetures constituent de véritables drames. Nos petites communes souffrent déjà d’une baisse démographique et du vieillissement de leur population ; la disparition des emplois industriels contribue à l’accélération de ces dynamiques négatives.

un accompagnement technique et financier important est nécessaire pour que ces initiatives soient couronnées de succès. Il est difficile de faire le tour de cette question cruciale en deux minutes, madame la secrétaire d’État. Aussi, j’aurais plaisir à vous accueillir dans mon département pour échanger davantage sur le sujet et approfondir la question.

que vous avez évoquées. Avant toute chose, je veux vous assurer qu’avec mes collègues du Gouvernement, Antoine Armand et Marc Ferracci, nous sommes aux côtés des salariés, de leurs représentants et des élus locaux pour réunir toutes les parties prenantes autour de la table, trouver des compromis et identifier des solutions pour préserver les sites et les emplois.

l’État s’est attaché, avec les partenaires locaux, à favoriser des reprises, avec des succès notables. C’est notamment le cas de la reprise par une Scop, qui vient d’être validée, de Bergère de France.

que les projets de reprise par des investisseurs reposent sur une vision industrielle pérenne et une stratégie de moyen ou long terme. Vous avez parfaitement raison de le souligner, madame la sénatrice, il s’agit d’un enjeu fondamental pour que les entreprises d’un territoire comme le vôtre puissent se développer structurellement sans être soumises à des stratégies d’investissement agressives. Je termine en vous assurant de l’attention du Gouvernement sur ces sujets, qui sont, vous l’avez également souligné, de véritables enjeux d’aménagement du territoire, notamment pour notre ruralité. La parole

Cet AMI visait à accompagner les territoires touchés par des restructurations économiques : 54 projets industriels pour un potentiel de 110 millions d’euros et la création de 300 emplois. L’agglomération de Morlaix a été retenue en décembre 2022 parmi les neuf territoires concernés au niveau national.

une phase d’investissement sur douze à dix huit mois, mobilisant une enveloppe de crédits de 1,5 million d’euros de soutien à l’investissement productif dédiée au financement de projets industriels innovants et structurants pour le territoire. Un comité de pilotage a eu lieu de janvier à avril 2023 afin d’identifier les projets innovants et les structures porteuses. L’idée était d’aller vite pour provoquer un choc industriel. Les dossiers priorisés et validés par le comité de pilotage territorial dans le cadre du dispositif « Rebond industriel » devaient être soumis au comité de pilotage ministériel opérationnel, placé auprès du Premier ministre, pour examen lors d’une réunion le 4 octobre 2023. Nous sommes en octobre 2024 et le choc industriel prévu n’est pas arrivé. En effet, seules deux entreprises ont été financées, à hauteur de 340 000 euros. Trois entreprises qui avaient prévu leur investissement ne sont aujourd’hui pas financées : Hemarina, entreprise innovante agissant dans la transplantation d’organes ; Sermeta, entreprise industrielle phare du pays de Morlaix ; et Ineo défense. Ma question est simple ces entreprises sélectionnées sur le territoire disposeront elles des sommes « levier » nécessaires à leurs investissements, et, si tel n’est pas le cas, que deviendront les fonds non utilisés fléchés pour les entreprises du pays de Morlaix ?

le territoire de Morlaix Communauté a en effet été lauréat de la première vague de l’AMI « Rebond industriel ». La phase d’ingénierie a permis, vous l’avez rappelé, d’identifier 54 projets. En complément des moyens d’ingénierie, le dispositif sanctuarise des crédits qui visent à soutenir des projets participant à la dynamique de rebond et de diversification du tissu industriel de ce territoire. Les projets recherchés par l’AMI sont donc des projets matures, avec un fort impact territorial, environnemental et sociétal.

Les deux entreprises ont signé leur contrat de subvention avec Bpifrance en décembre 2023. Je vais maintenant vous répondre sur les trois autres entreprises que vous avez évoquées et qui se sont vu notifier un refus. refus. Le projet de l’entreprise Ineo Défense n’a pas pu faire l’objet d’un soutien, compte tenu du droit européen en matière d’aides d’État. S’agissant du projet Sermeta, qui visait à soutenir l’industrialisation de pièces pour chaudières à gaz, il entrait en contradiction avec les objectifs de planification écologique du Gouvernement. Enfin, pour le projet de l’entreprise Hemarina, l’Agence de l’innovation en santé (AIS) n’a pas considéré les essais cliniques suffisamment probants.

Monsieur le président, madame la ministre, dans le Sud Grenoblois, tout un écosystème industriel pourrait disparaître si l’usine Vencorex n’était pas reprise. Fragilisée par la concurrence chinoise et placée en redressement judiciaire, cette entreprise est au cœur de la chimie locale. Avec sa voisine Arkema, dont l’État est actionnaire, elle produit du chlore, de l’eau oxygénée, des tolonates – des composants pour peintures et vernis – et du perchlorate, un élément du carburant de la fusée Ariane. Avec le chlore, Framatome produit notamment des éponges de zirconium pour le gainage des réacteurs nucléaires. La fermeture de Vencorex aurait donc des conséquences en cascade catastrophiques. Toujours en Isère, le fabricant de panneaux solaires Photowatt, essentiel pour la transition énergétique, est en train de mourir du dumping étranger, notamment chinois, comme GE Hydro voilà quelques années. En Savoie, une usine Ferroglobe produisant du silicium a fermé en 2022 et le site de Niche Fused Alumina (NFA), qui produit de l’alumine et du corindon blanc, indispensables à des usages de pointe, a failli être liquidé. À chaque fois, les plans sociaux s’enchaînent et un riche savoir faire s’éteint. Depuis la pandémie, qui nous a rappelé combien la dépendance à l’égard de pays étrangers posait problème, le Gouvernement ne cesse de parler de souveraineté industrielle, mais les actes ne suivent pas. Face à la mondialisation débridée, l’État reste trop souvent attentiste. Salariés et élus locaux ne cessent pourtant de vous interpeller, ainsi que le Premier ministre, sur les conséquences de ces fermetures pour l’emploi, pour la balance commerciale et pour notre souveraineté. Quels moyens l’État se donne t il pour faire pression sur les grands groupes, dont il est parfois actionnaire ?

en matière de défense de nos industries stratégiques. Concernant tout d’abord l’accompagnement des entreprises fragiles, avec mes collègues Antoine Armand et Marc Ferracci, nous sommes aux côtés des salariés, de leurs représentants et des élus locaux pour, dans chacune des situations, mettre toutes les parties prenantes autour de la table

alors que l’entreprise était en redressement judiciaire. Vous avez cité également l’usine Vencorex au Pont de Claix, en Isère. Cette entreprise du secteur de la chimie est actuellement en redressement judiciaire. Marc Ferracci et ses équipes sont en lien permanent avec les organisations syndicales, la direction et les élus. Le ministre porte une attention particulière au devenir des salariés et, plus largement, à la pérennité de la plateforme du Pont de Claix, aussi bien pour des enjeux environnementaux que de sécurité. Au delà de ces cas particuliers, notre action vise à défendre des mesures structurelles pour nos industries stratégiques. Nous sommes bien conscients, monsieur le président Gontard, des fragilités de certaines filières,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, par le nombre de ses victimes – 100 000 à l’horizon 2025 –, l’amiante constitue un scandale sanitaire historique qui n’a pas fini de faire parler de lui. Devant nous est ouvert l’immense chantier du désamiantage et du traitement des déchets, véritable enjeu de santé publique et de sécurité sanitaire

Quelques solutions alternatives sont en cours de développement ou existent déjà, notamment l’inertage par vitrification, qui détruit totalement l’amiante. Dès 2014, un rapport sénatorial sénatorial préconisait la mise en place d’une structure interministérielle chargée d’une coordination publique. Allant plus loin dans le même esprit, des associations de victimes proposaient la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante regroupant acteurs publics et privés de la filière du désamiantage. La feuille de route pour le traitement des déchets d’amiante, censée éviter leur stockage et qui avait été inscrite dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, était attendue pour 2023. Elle n’a toujours pas été rendue publique et il semble qu’aucun projet ne soit soit en cours pour imaginer, tester et développer au niveau adéquat des méthodes alternatives à l’enfouissement. J’ajoute que cette inaction, couplée aux coûts importants demandés par les entreprises spécialisées pour démonter et évacuer les déchets, conduit à des comportements inadaptés et dangereux, avec notamment des dépôts sauvages dans l’espace public public de déchets hautement toxiques. Ma question est donc double, madame la secrétaire d’État : quelles suites comptez vous donner aux différentes préconisations émises depuis dix ans en matière de recyclage des déchets d’amiante ? Pouvez vous préciser les intentions du Gouvernement,

Pour en améliorer la collecte, la loi antigaspillage de 2020 est venue renforcer les moyens d’action du maire et les sanctions contre les responsables de dépôts sauvages de déchets. Cette loi a également conduit à la mise en place, en 2023, de la filière à responsabilité élargie

cette technique, bien que ne permettant pas de détruire les fibres d’amiante, constitue un moyen sûr de traiter ces substances en permettant d’éviter leur dispersion dans l’environnement. Pour autant, madame la sénatrice, les solutions alternatives à l’enfouissement font l’objet d’une attention particulière en France.

En 2009, les pays les plus riches ont accepté de mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement afin de les aider à s’adapter au changement climatique. Un nouvel objectif de financement devrait être formalisé lors de la COP29. C’est dire l’importance de ce rendez vous. Mais pourquoi à Bakou, en Azerbaïdjan,

notoire au régime, réfugié sur le territoire français. Qui plus est, cet État mène des opérations hostiles contre la France en Nouvelle Calédonie, en nous traitant de colonisateurs. L’Azerbaïdjan n’est pas une grande puissance militaire, mais c’est une puissance d’influence malveillante qui ne se prive pas d’attaquer fortement la France. Enfin, ce pays

t elle à cette occasion un message fort à l’encontre de ce régime qui porte atteinte aux droits de l’homme et qui met en cause la liberté dans l’ensemble de la région ? La secrétaire d’État. Madame la sénatrice Carlotti, fin 2023, les Nations unies ont choisi l’Azerbaïdjan pour présider la COP29 en fonction de leurs propres règles et en suivant le principe de rotation géographique. L’Azerbaïdjan a été choisi par consensus par par le groupe Europe de l’Est, l’un des cinq groupes géographiques de l’ONU. La France, fidèle à son engagement climatique et à l’héritage de l’accord de Paris de décembre 2015, reste pleinement engagée dans les négociations climatiques. C’est pourquoi la ministre Agnès Pannier Runacher se rendra à Bakou à Bakou pour la COP29. Les enjeux de cette COP sont importants. Il s’agit de trouver un accord sur le nouvel objectif collectif quantifié sur la finance climat mondiale, qui doit succéder à l’objectif de 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025. Il s’agira aussi d’étudier l’article 6 sur les marchés carbone afin de définir un cadre international sur ce sujet. Il faudra, enfin, travailler à l’atténuation, notamment pour définir le cadre des futures contributions nationales que chaque pays doit présenter d’ici au mois de février 2025 pour actualiser son programme de baisse d’émissions et respecter la trajectoire de 1,5 degré. Pour autant, madame la sénatrice, les droits de l’homme sont toujours au cœur de notre diplomatie, conduite par mon collègue Jean Noël Barrot sous l’autorité du Président de la République. Nous serons donc très vigilants sur la participation de la société civile et sur le respect de ses droits lors de cette COP29. Nous avons d’ailleurs déjà fait passer des messages dans ce sens à la présidence de l’Azerbaïdjan, qui est tenue de respecter les règles des Nations unies à cet égard. La parole est à Mme

Monsieur le président, madame la ministre, l’eau que nous buvons est massivement contaminée par un polluant éternel, l’acide trifluoroacétique, autrement nommé TFA. Cette contamination a été révélée cet été par plusieurs rapports du Réseau européen d’action sur les pesticides et de l’association Générations Futures. Selon ces travaux, 100 % des eaux de surface et souterraines testées sont contaminées. Pire, 94 % des eaux du robinet sont, elles aussi, contaminées.

avec une moyenne de 2 100 nanogrammes par litre. Il n’y a là rien de surprenant quand on sait que les zones de captage de l’eau potable ne sont protégées ni de l’épandage de pesticides, probablement responsable de la présence de TFA, ni des forages pétroliers, responsables de la pollution aux hydrocarbures de l’eau, comme à

participer à cet effort. Le plus alarmant reste évidemment l’absence de surveillance toxicologique de ces composés chimiques, et ce malgré les alertes des scientifiques.

ministre, alors que l’Allemagne a récemment demandé de classer le TFA comme substance reprotoxique ? Nous devons faire preuve d’autant plus de précautions que le caractère éternel de ce polluant a pour conséquence une accumulation inéluctable dans l’eau tant que les sources de ce métabolite sont utilisées et répandues dans l’environnement. Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement va t il se se saisir de la question de la pollution au TFA ?

Les éléments de l’Anses font partie intégrante du plan d’action interministériel sur les PFAS publié en avril 2024. Ce plan s’attache, dans un objectif de prévention, à réduire les émissions de PFAS, la contamination des milieux, ainsi que l’exposition des populations et des et des écosystèmes. Concernant plus spécifiquement le TFA, sachez que la présence de cette substance est mesurée dans les eaux dans le cadre de la campagne nationale exploratoire mise en œuvre par le laboratoire d’hydrologie de Nancy sur la période 2024 2026. La Commission européenne a demandé à l’Allemagne de soumettre un dossier de classification pour le TFA à l’Agence européenne des produits chimiques en mars 2024. L’issue de ces travaux sur les dangers de ce métabolite permettra d’éclairer la question.

pour qu’elle fixe les valeurs toxicologiques de référence pour le TFA. Les conclusions de ces travaux sont attendues pour fin octobre 2025. Elles contribueront à déterminer les valeurs de gestion dans les différents milieux, dont les eaux,

Ce dispositif est issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi Agec, qui avait pour ambition, notamment, « de favoriser les produits les meilleurs pour l’environnement et de permettre de réduire le prix des produits vertueux Or nous constatons que les textes réglementaires d’application qui se sont succédé depuis 2020 produisent des effets inverses et pénalisent dangereusement les produits qui stockent du carbone – je pense en particulier au bois à l’encontre même des objectifs de décarbonation pourtant reconnus encore récemment comme prioritaires, et notamment dans le bâtiment, avec la réglementation environnementale (RE) 2020. Selon les estimations de la Fédération nationale du bois, l’écocontribution

regard des très importantes distorsions de concurrence que pourraient induire ces décisions qui ne reconnaissent pas suffisamment les propriétés écologiques du bois. Plusieurs éco organismes ont même décidé de geler les hausses prévues de cette contribution financière que versent les entreprises. La filière pourrait en effet se retrouver grandement fragilisée si rien n’est fait pour corriger ces contradictions.

La mise en place de cette filière, vous le savez, était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités locales, qui supportent aujourd’hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment et font face au phénomène des dépôts sauvages. En ce qui concerne le cas particulier du bois, le Gouvernement est attentif à la situation économique de ce secteur. Ainsi, plusieurs mesures ont d’ores et déjà été prises pour permettre de diminuer l’enveloppe globale des coûts supportés pour le bois. Des arrêtés ont ainsi été récemment publiés pour contraindre les éco organismes à faire évoluer la structure du barème d’écocontribution bois, afin qu’elle soit différenciée entre les produits en bois frais, d’une part, et les produits bois secs et rabotés, majoritairement importés, ce qui constitue une première avancée face au risque de distorsion de concurrence que vous évoquez. Il est également imposé aux éco organismes de prévoir un abattement de contribution pour les produits générant des déchets parmi les mieux valorisés, ce qui va également favoriser le bois. Le gain pour la filière est estimé à près de 45 millions d’euros. Par ailleurs, un projet de décret est en cours de validation, qui permettra de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches. Cela devrait permettre un gain pour l’ensemble de la filière REP d’au moins 180 millions d’euros. Enfin, les éco organismes ont commencé à mettre en place des primes pour les produits intégrant des matériaux issus de ressources renouvelables gérées durablement et ont été incités à amplifier ces primes, ce qui devrait également profiter à la filière bois. La parole

budgétaire. Un rapport du Sénat a déjà montré que l’enveloppe allouée aux travaux nécessaires pour les casernes était systématiquement inférieure de 50 % aux besoins d’investissement. Les collectivités, mais aussi les bailleurs,

que les loyers versés n’étaient pas ajustés en fonction de l’évolution des taux d’intérêt des emprunts contractés pour financer la construction du casernement. Le déséquilibre financier s’élèverait ainsi à 35 000 euros pour l’exercice 2024. Loin des déclarations laissant entendre que les collectivités contribueraient au déficit du pays, on voit bien au contraire qu’elles investissent et qu’elles contractent des emprunts pour garantir les

Dans l’attente, la tension qui pèse sur la trésorerie de la gendarmerie a conduit à donner la priorité au financement des activités opérationnelles, pour permettre la poursuite de l’engagement des unités de gendarmerie au service de la sécurisation du territoire national. Aussi, outre le report de certains investissements, la mise en paiement de certains loyers a été retardée. La mesure porte sur le report des seuls loyers de septembre, octobre et novembre souscrits auprès de bailleurs institutionnels métropolitains, collectivités ou sociétés anonymes. Les baux faisant l’objet d’un report de paiement représentent un montant total de 90 millions d’euros. Les bailleurs les plus fragiles, notamment les particuliers, ne sont pas concernés, de même que l’ensemble des bailleurs des outre mer. Par ailleurs, pour permettre aux bailleurs concernés de signaler les difficultés particulières auxquelles cette mesure pourrait les exposer, une procédure de recensement des baux devant faire l’objet d’une mesure d’exception a été mise en place par le ministre de l’intérieur, en lien avec les directions départementales des finances publiques. Dans tous les cas, le ministère de l’intérieur s’engage à procéder au règlement des loyers et des intérêts moratoires associés courant décembre, dès lors que les crédits supplémentaires sollicités auront été débloqués. De manière plus globale, le ministre de l’intérieur souhaite conduire une réflexion de fond sur le devenir du modèle immobilier de la gendarmerie. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit notamment de reprendre l’entretien du parc domanial. Je m’associe enfin à vos propos : en tant qu’élu local, je sais bien qu’en France les collectivités contribuent à l’investissement et non au déficit.

de plus en plus souvent au péril de leur intégrité physique, viennent de signer, avec le préfet du département, un protocole relatif au traitement des infractions et atteintes faites aux élus dans le ressort de la cour d’appel de Metz. Ce texte, qui vise à améliorer la lutte contre les violences et autres atteintes faites aux maires, à leurs adjoints et aux élus en général, pour que force reste à la loi, réunit la Fédération des maires de Moselle, l’Association des maires ruraux

Il associe ainsi tous les échelons institutionnels directement concernés par cette problématique. Aussi, pour que cette union des forces soit couronnée de succès, il conviendrait d’en faire la promotion une campagne dans les médias qui viendrait affirmer et appuyer la volonté intraitable de l’État de mettre un terme à des comportements et des actes inadmissibles dans nos sociétés, où le vivre ensemble implique le respect de la loi et de ses représentants.

et la protection des maires et des élus locaux. Il faut l’utiliser pleinement ! Pour ce qui concerne le ministère de l’intérieur, la vigilance et la mobilisation sont au rendez vous. Comme vous le savez, un Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (Calaé) a été créé en mai 2023 et un certain nombre de dispositifs opérationnels ont été mis en œuvre,

Collectivement, nous ne devons laisser passer aucune de ces dérives honteuses. Je vous remercie, monsieur le sénateur, d’avoir évoqué l’exemple très concret du protocole extrêmement utile qui a été signé à Metz. Vous pouvez compter sur le soutien et sur la détermination du Gouvernement.

ont dressé un constat inquiétant sur la médecine scolaire et la santé à l’école. Ce constat doit nous inciter à réagir rapidement. La santé psychologique de nos jeunes, vous le savez, ne cesse de se dégrader, au point que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale en 2025. Les médecins titulaires et contractuels en activité sont trop peu nombreux. La démographie médicale a fortement décru entre 2017 et 2021, et les départs à la retraite vont s’accélérer dans les deux prochaines années. Dans le département de l’Essonne, la situation n’est guère reluisante, avec un peu moins de 14 postes en équivalent temps plein (ETP) pourvus sur 36, alors que le nombre d’élèves à prendre en charge ne cesse d’augmenter ! Plusieurs enjeux doivent Comment garder les médecins titulaires à leur poste ? Il est urgent, selon moi, de réévaluer leur grille indiciaire et de redéfinir rapidement des missions et des objectifs de santé qui ont du sens et qui sont réalisables. Comment attirer de nouveaux médecins contractuels ? Un salaire attractif est indispensable ; il doit être cohérent avec celui des médecins titulaires en début de carrière. Comment revaloriser un métier que les médecins scolaires exercent dans des conditions matérielles de plus en plus précaires, sans locaux, sans moyens pour les dépistages, sans accès partagé aux données de santé, sans véhicule pour les déplacements, sans assistante médicale ? Comment assurer une meilleure coordination avec les autres professionnels de santé, au plus près des usagers ? Comment, enfin, mieux associer les médecins scolaires au processus de décision des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre de la scolarisation inclusive ? Dans ce contexte bien sombre, il est urgent d’agir. Aussi, monsieur le ministre, ma question est la suivante : quelles initiatives fortes entendez vous prendre dans les prochaines semaines pour revaloriser la médecine scolaire et répondre aux besoins de santé grandissants des élèves ? La parole

Comme vous le savez, afin de renforcer l’attractivité du métier d’infirmière scolaire, le ministère a revalorisé leur rémunération, en mai dernier, à hauteur de 200 euros net par mois. Par ailleurs, pour répondre aux difficultés que vous avez très justement soulevées,

pour assurer le relais des diagnostics des médecins scolaires. Je compte sur vous pour mener à bien une réflexion interministérielle sur ce sujet très important, conformément à ce que vous venez d’annoncer.

Au mois de janvier 2024, les représentants de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) de Mayotte m’ont indiqué, à l’occasion d’un entretien, que près de 20 000 enfants sont actuellement non scolarisés à Mayotte. Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous m’indiquiez si ces chiffres sont exacts.

À la rentrée 2024, 63 800 élèves sont scolarisés à Mayotte dans le premier degré, soit un millier de plus qu’à la rentrée précédente. Pour faire face à ces besoins, 1 063 emplois d’enseignants ont été créés dans le premier degré depuis 2018, ce qui a permis d’absorber le flux et même de rattraper le retard. entre 2019 et 2023, le taux de scolarisation à l’âge de 5 ans est passé de 85 % à 95 %, ce qui représente une nette amélioration. Si les emplois et la solidarité nationale sont au rendez vous,

Dans le même temps, nous renforçons les moyens du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (Casnav). Toutefois, tous les enfants présents sur le territoire ne sont pas connus

Madame la ministre, je souhaite vous interpeller au sujet de la situation incompréhensible que subit le plan Destination France. Destiné à une relance du tourisme, ce plan a été annoncé, à grand renfort de communication, par le gouvernement démissionnaire. La mesure « Ports de plaisance d’avenir » a officialisé un engagement pris par l’État, à hauteur de 20 millions d’euros, au travers d’un dispositif opéré par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Des appels à projets ont été lancés afin de sélectionner les meilleures candidatures et de soutenir des actions structurantes pour les territoires. Cette mesure, de même que les projets et les lauréats, ont fait l’objet d’annonces et de notifications officielles publiées par le précédent gouvernement.

Cette situation suscite beaucoup d’incompréhension et d’inquiétude parmi les acteurs de la filière touristique nautique, qui se retrouvent ainsi soudainement mis en difficulté. Au delà du fait que cette situation décrédibilise la parole de l’État, certaines opérations déjà engagées pourraient être remises en cause ou subir un surcoût pour les maîtres d’ouvrage.

cette incertitude concernant les crédits et des difficultés qu’il avait à confirmer le versement des subventions demandées. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que cette situation génère pour des projets qui ont été engagés.

en faveur de chacun de ces projets. Des discussions sont en cours pour lever ces difficultés, ce qui permettrait de confirmer tout ou partie des subventions

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Mickaël Vallet, votre question porte sur une filière économique extrêmement importante, l’ostréiculture et la conchyliculture.

du norovirus de l’hiver 2023 2024. Il a en effet activé des mesures de trésorerie, mais aussi de communication. Ainsi, 500 000 euros ont été mis sur la table dans le cadre du dispositif « communication de crise

a également débloqué des fonds pour accompagner l’équipement en bassins de purification le fonds pour la transition écologique.

Si, à l’issue de ce projet, au mois de décembre 2025 – voilà un calendrier précis –, la méthode se révélait convaincante, cette technique pourrait être reconnue et mobilisée dans l’ensemble du territoire, après évolution de la réglementation européenne.

à l’abri tout ou partie de la production, notamment à l’occasion des pics de consommation, essentiels pour cette activité économique. Le Gouvernement vise, à terme, l’amélioration structurelle de la qualité de l’environnement dans lequel les professionnels travaillent.

Nombre d’entre elles connaissent des difficultés pour s’assurer et déplorent une dégradation de leurs relations contractuelles avec les assureurs. Cette dégradation se traduit par des ruptures unilatérales et brutales de contrats, des hausses de tarifs, des primes et des franchises, voire l’absence de réponse des assureurs aux appels d’offres publiés par les collectivités. Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle s’aggrave.

un problème important dans leur relation avec leur assureur ; ce taux s’élève à 90 % pour les collectivités de plus de 10 000 habitants. Étonnamment, les résiliations unilatérales et la hausse des prix subies par les collectivités ne sont pas directement liées à une augmentation de la sinistralité. En réalité, elles révèlent une véritable instabilité des contrats et les dysfonctionnements du marché de l’assurance, notamment un phénomène de concentration sur le marché de l’assurance, un oligopole qui prive de choix les collectivités et les soumet aux seules décisions de quelques acteurs. Incontestablement, le manque de concurrence entre les assurances amène les collectivités à se soumettre à ces hausses de tarifs. Face aux relations particulièrement dégradées et déséquilibrées entre les collectivités et les assureurs, qu’envisagez vous,

qui méritent d’être corrigés dans le contexte économique particulièrement difficile que nous connaissons. La modification du seuil de tension de la demande de logements sociaux imposée par le décret du 29 mars 2023

conséquence d’une obligation qu’elles ignoraient pourtant jusqu’alors ! Dans le même ordre d’idée, est il normal d’infliger une pénalité pour non atteinte des objectifs de production de logements sociaux

leur échappent. Déjà fragilisées par un contexte économique complexe, elles voient leurs efforts pour construire des logements sociaux méprisés, malgré les réalités locales qu’elles doivent affronter

de nombre de ponts et mettre en exergue les lourdes conséquences induites pour les communes concernées, qui doivent prendre des mesures restreignant la circulation et se trouvent limitées dans leur capacité financière.

Aussi, quelles mesures le Gouvernement compte t il mettre en place sans que cela obère les canaux de financement traditionnellement usités par les communes pour d’autres projets importants ? dans la proposition n° 2 du rapport sénatorial d’information sur la sécurité des ponts la constitution d’un fonds pérenne pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l’entretien et la réparation de leurs ouvrages d’art. Peut on y donner suite ? ministre, compte tenu de la fin programmée du programme national Ponts en 2025, envisagez vous de mettre en place un nouveau programme ? Pourquoi ne pas prévoir des crédits dans les futurs contrats de plans et fonds structurels européens ? Excellente

80 000 dossiers de pénalités et 600 000 « courriers pédagogiques » envoyés par le concessionnaire. C’est dire l’incompréhension des utilisateurs ! En pratique, l’absence de portail de télépéage de télépéage induit en erreur et laisse à penser que ce tronçon est gratuit. Pour les détenteurs d’un badge de télépéage, l’opération se révèle indolore, leur compte étant automatiquement prélevé.

continue du paiement spontané. Le principe de la plateforme de paiement internet unique est d’ores et déjà intégré au nouveau cahier des charges type des contrats de concession. Pendant les premiers mois d’exploitation, les sociétés permettent aux usagers qui se trouvent pour la première fois en dépôt de paiement de régler leur péage sans majoration dans des délais suffisants.

et les nuisances liées au chantier. Ce projet d’intérêt national est pourtant vital à bien des égards pour la Normandie, en particulier pour le Calvados. Tous deux pâtissent en effet depuis trop longtemps d’une mauvaise desserte ferroviaire frappant le transport tant de voyageurs – les usagers de la ligne Paris Cherbourg au quotidien que de marchandises. Annoncé par Nicolas Sarkozy en 2009, ce projet largement transpartisan a depuis été défendu par les présidences successives de François Hollande et d’Emmanuel Macron. Son aspect prioritaire a été confirmé à maintes reprises par la commission Mobilité 21 et le Conseil d’orientation des infrastructures (COI). Qui plus est, on ne compte plus le nombre de ministres ayant reconnu la dette ferroviaire de l’État à l’égard de la Normandie. Aujourd’hui, l’enjeu de la LNPN réside surtout dans l’amélioration structurelle de la fiabilité de la ligne et l’augmentation de sa capacité, en l’état impossible du fait de sa saturation.

de gaz à effet de serre. La LNPN doit favoriser le désenclavement de la Normandie, un territoire stratégique qu’il convient de relier efficacement à Paris et à l’ensemble du pays. Il ne s’agit pas d’un simple projet ferroviaire, mais bien d’un levier incontournable de compétitivité, de modernisation et de développement durable, au service de la croissance dans des départements comme le Calvados et, plus largement, pour la France. Avec l’aménagement de la vallée de la Seine, c’est aussi une partie de la politique maritime du pays qui se joue. Pour toutes ces raisons, je vous demande, madame la ministre, de réaffirmer l’engagement total de l’État dans ce projet essentiel, qui doit être mis au rang des priorités du Gouvernement. La parole

et donc de la Normandie, tout en respectant naturellement les préoccupations de chacun d’entre eux. C’est dans ces conditions que seront envisagées dans les toutes prochaines semaines

Alors que l’État a déjà mis fin, sous les précédents gouvernements, au projet de l’autoroute A45, pour lequel 400 millions d’euros sont budgétés en substitution, il conviendrait que les habitants de la métropole de Saint Étienne ne subissent pas une double peine.

apporter pour fluidifier les déplacements et respecter ses engagements concernant des équipements d’envergure et structurants, comme cet échangeur de la Varizelle à Saint Chamond

dit de la Varizelle, dans le département de la Loire. Cette opération s’inscrit, en effet, dans le programme multimodal d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint Étienne,

près de 190 millions d’euros auront été mobilisés, dont plus de 70 % pour le volet ferroviaire et 30 % pour les autres Nul ne conteste au sein du Gouvernement la nécessité de respecter les engagements de l’État, notamment en complétant l’actuel demi échangeur de la Varizelle pour améliorer la fluidité, mais aussi sécuriser les transports. L’État, qui est le maître d’ouvrage de ce projet,

De ce fait, il génère de fortes nuisances sanitaires et environnementales, dont il a été montré qu’elles pouvaient entraîner la perte de trois ans de vie en bonne santé pour les riverains.

C’est sur le fondement de ces conclusions que les ministres ont soumis à la consultation du public, du 29 avril au 29 juillet, un scénario conjointement sélectionné,

je vais vous parler d’un sujet qui vous est cher. Alors que va s’ouvrir dans quelques jours le congrès des maires et des élus locaux, aurez vous une bonne nouvelle à leur annoncer ? Ce sont eux qui gèrent au quotidien ces mini républiques que sont les communes. Ils se dépensent sans compter, donnant leur énergie et leur temps. Ces élus de proximité sont la première porte pour la solidarité nationale. Et nous savons combien il est difficile de concilier

le régime social, la formation et la reconversion, la responsabilité pénale et la déontologie des élus. Dans mon département, une femme maire a été gravement insultée et menacée de mort.

Le Premier ministre a confirmé son intention de faire prospérer le débat et d’aboutir à ce que j’appelle un statut, en tout cas à des dispositions favorables à l’engagement citoyen.

avec peu. Je souhaite donc vous interroger sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), essentielle à nos territoires et dont le sort me paraît incertain. Les plafonds de dépenses prévisionnelles de la loi de finances pour 2025 prévoient un montant de DGF identique à celui de 2024, soit 27,2 milliards d’euros. Or les compétences déléguées par l’État aux collectivités territoriales augmentent d’une année sur l’autre, ce qui alourdit leurs charges de fonctionnement et limite leurs capacités d’investissement. Cette situation de déséquilibre est un sujet d’inquiétude pour les élus. Le désengagement de l’État depuis une décennie est indéniable. Entre 2014 et 2017, la DGF a été réduite de 10 milliards d’euros. Entre 2018 et 2022, son montant a stagné pour se fixer aux alentours de 27 milliards d’euros. Pèsent aussi sur les comptes des collectivités : la suppression de la réserve parlementaire en 2017 et de la taxe d’habitation en 2023 ; l’explosion du coût de l’énergie et l’augmentation de la masse salariale ; la réduction du fonds de compensation pour

particulièrement pour nos communes rurales, qui sont les premières victimes de cette politique consistant à déléguer toujours plus et financer toujours moins. Le Premier ministre assurait pourtant, ici même, qu’il travaillerait avec les collectivités territoriales : « pas sans elles, pas contre elles

requiert absolument un redressement qui, naturellement, génère une contraction budgétaire, c’est à dire de vraies difficultés. Il appartiendra au Parlement

Ma question porte sur les sites internet frauduleux, dont l’interdiction ferait faire des économies à l’État, et dont personne ne regretterait la disparition.

Les promesses de ces sites sont malheureusement à la hauteur des espérances des patients les moins citoyens : taux d’acceptation des arrêts de 100 %, arrêt garanti et accepté en moins de cinq minutes.

J’ai déjà interpellé plusieurs ministres sur le sujet, et je l’ai soulevé il y a plus de dix jours lors d’une audition. Ce matin, ces sites internet étaient encore en ligne. Je ne donnerai pas leurs noms pour ne pas leur faire de publicité, mais je les tiens bien évidemment à votre disposition.

je souhaite tout d’abord vous remercier pour votre engagement contre cette dérive inadmissible et que nous devons combattre : l’existence de sites qui délivrent de manière frauduleuse des arrêts de travail. En 2023, les faux arrêts de travail ont constitué un préjudice de 7,7 millions d’euros pour l’assurance maladie, contre 5 millions d’euros Nous devons donc lutter contre ces pratiques frauduleuses. La Cnam a engagé plusieurs actions pour détecter les arrêts de travail falsifiés et les empêcher. Il s’agit de lutter contre les fausses déclarations sociales d’indemnités journalières et de mieux identifier les faux déclarants. En 2023, plus de 1 million de contrôles ont été menés par le service médical de la Cnam sur les arrêts de travail en cours et plus de 77 000 reprises de travail ont été notifiées.

a signalé plusieurs sites au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Il appartient dorénavant aux juridictions de conduire les enquêtes et de réprimer ces fraudes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, La mortalité infantile a augmenté fortement en France au cours des dernières années. Le constat est sans appel : en 2023, on aura atteint un seuil de 4 décès pour 1 000 naissances, soit le taux le plus élevé depuis vingt ans.

des handicaps d’origine périnatale. On observe que la mortalité infantile est beaucoup plus forte dans les départements les plus pauvres et les plus ruraux. Les causes, vous les connaissez : fermetures de lits, difficultés d’accès aux soins, pénurie de soignants, fermeture des services, insuffisance du nombre des maternités.

de tomber enceintes afin d’éviter tout drame ? Madame la ministre déléguée, ma question est simple : comment faire pour réarmer démographiquement la France et sauver des vies sans moyens humains, matériels, financiers ?

je vous remercie pour votre question et je partage vos constats sur la situation de la périnatalité en France. Depuis quelques années, le taux de mortinatalité spontanée et de mortalité infantile stagne, voire se dégrade. Nous ne pouvons évidemment pas nous en contenter.

de réanimation néonatale pour 1 000 naissances dans chaque région d’ici à 2027. Et 600 postes d’internes seront proposés chaque année en pédiatrie, soit une augmentation de 75 % par rapport à 2022. Cette feuille de route prévoit aussi un travail de collecte sur les données de santé, en complément des mesures existantes pour améliorer la qualité des données périnatales. Les certificats de décès néonataux ont été étendus de l’âge de 28 jours à 1 an de l’enfant, et des travaux d’analyse en cas de décès des nouveau nés à terme ou à proximité du terme ont été lancés en 2023. Les premiers résultats sont attendus d’ici à la fin de l’année. voulons faire de la prévention une priorité pour la santé périnatale, notamment par la démarche du « aller vers » les populations les plus éloignées du système de santé,

Enfin, le Gouvernement continue de porter une grande attention aux fermetures de maternité. Lorsqu’une fermeture s’impose pour ne pas faire peser de surrisques sur la mère et l’enfant, la priorité est donnée au maintien

Ce n’est pas la bonne manière de traiter la question. Il faut revoir le maillage des maternités, sachant qu’un trajet de quarante cinq minutes pour accéder à une maternité double le taux de morbidité tant pour la mère que pour que pour l’enfant. Enfin, des postes d’internes doivent être ouverts aux futurs médecins, même à ceux ayant étudié à l’étranger, qui doivent être affectés en France dans les établissements en tension. Des médecins français étudient

Cela a une incidence sur le désengagement par les services de prévention et de santé au travail du suivi des agents de la fonction publique. De plus, cela interroge quant à l’efficacité et à la pérennité de la protection de la santé des travailleurs dans ce secteur.

Cette situation préoccupante est illustrée de manière frappante dans la Sarthe, où l’association Santé au travail 72 a dû prendre la décision radicale d’arrêter le suivi en santé au travail des collectivités et des établissements qu’ils accompagnaient jusqu’alors. telle décision frappe directement les 10 000 agents, les laissant sans le soutien médical et préventif nécessaire à leur bien être au travail. La réforme visait initialement à moderniser et à renforcer le système de santé au travail. Mais son application a révélé des failles importantes dans la planification et la gestion des ressources. Les services de santé au travail se retrouvent débordés, incapables de faire face à la demande croissante de suivi médical et de prévention. En l’absence de suivi médical régulier, les agents sont exposés à des risques accrus de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

Aussi, pouvez vous m’indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement compte prendre pour faire face à la pénurie de médecins au travail, tout en garantissant que les services de prévention et de santé au travail disposent des ressources nécessaires pour accomplir leurs missions ? La parole

impose aux autorités territoriales de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents. Les missions de cette médecine préventive sont assurées par une équipe pluridisciplinaire, dont un médecin du travail, qui peut appartenir au au service créé par la collectivité ou l’établissement, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; il peut encore relever directement des administrations lorsque celles ci disposent des moyens nécessaires. À titre subsidiaire, les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) peuvent être sollicités s’ils disposent des ressources suffisantes pour assurer le suivi médical des agents publics. Lors d’une demande d’agrément, une Dreets peut demander à un SPSTI de cesser de suivre un public s’il ne dispose plus de la ressource médicale suffisante pour mener à bien ses missions prévues

par les centres de gestion de la fonction publique compétents localement pour les agents publics. La Dreets s’est par ailleurs engagée, aux côtés de l’agence régionale de santé (ARS), dans une procédure de recrutement de praticiens avec autorisation d’exercer, pour faciliter l’installation dans la région de quatre médecins du travail diplômés. La parole est

que sur la diminution de près de 30 % du budget alloué au centre de coordination des dépistages des cancers en Nouvelle Aquitaine. Il m’avait alors été répondu ceci : « La diminution des budgets qui lui sont alloués ne s’accompagnera pas d’une baisse de l’activité de dépistage. Elle est uniquement liée au transfert de certaines missions à l’assurance maladie, dont l’envoi de courriers. »

du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, des actions spécifiques d’« aller vers » ou encore le dépistage organisé du cancer colorectal. Au nom du principe d’égalité,

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Nicole Bonnefoy, vous m’interrogez sur les réductions budgétaires concernant le centre de prévention et de dépistage des cancers de Nouvelle Aquitaine, ainsi que sur l’impossibilité pour celui ci de remplir

Je demande sincèrement au Gouvernement de reconsidérer cette mesure budgétaire, qui est un non sens sanitaire et financier. Les équipes locales ont besoin d’être confortées dans leur mission, alors que leurs objectifs sont atteints. Entendez les ! Entendez les élus ! La parole

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, des référents handicap doivent être recrutés dans toutes les universités de France et se charger d’accompagner et d’aider les étudiants en situation de handicap. À la rentrée 2022, on dénombrait plus de 59 000 étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur, soit sept fois plus qu’il y a vingt ans. C’est une bonne chose, me direz vous. Néanmoins, le cheminement de ces étudiants dans l’enseignement supérieur demeure compliqué, voire très compliqué. D’après les chiffres diffusés par les services du ministère, un étudiant en situation de handicap sur cinq ne bénéficie encore d’aucun aménagement. Toujours d’après les chiffres fournis, les étudiants handicapés se concentrent en licence et deviennent moins nombreux au fil du cursus universitaire. Les remontées de terrain font apparaître que les référents handicap sont peu connus et manquent de formation. Ainsi, selon une étude menée pour le compte des huit fédérations d’étudiants dans le secteur de la santé, 44,5 % des sondés estiment que les référents handicap ne sont pas clairement identifiés,

depuis la loi du 11 février 2005. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Deux circulaires, du 6 février 2023 et du 10 juillet 2024, ont précisé le cadre des aménagements possibles pour les étudiants en situation de handicap dans leur parcours de formation et pour les examens et concours. En complément, une communication volontaire a été lancée pour aider les étudiants et les établissements les accompagnant. Ainsi, un guide vers l’autonomie a été adopté au mois d’octobre 2024 ; il donne des exemples de bonnes pratiques mutualisables dans les établissements universitaires. L’accès aux études supérieures est facilité financièrement dès l’entrée en cycle de licence grâce aux quatre points de charge supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap. Cet engagement vise l’ensemble du parcours, de Parcoursup jusqu’au plus haut niveau de formation.

Afin de les professionnaliser, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a établi deux modèles de fiches de poste définissant leurs missions et transmises aux établissements et il anime l’ensemble du réseau, en lien avec l’Association des qui regroupe les référents handicap. Le projet de loi de finances 2025 dote les établissements avec une enveloppe de 21 millions d’euros, soit une multiplication par trois en trois ans des

un agent âgé de 52 ans a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe après avoir été ébouillanté par un détenu. Je souhaite tout d’abord exprimer mon plein soutien au surveillant agressé et à ses collègues ; je comprends parfaitement leur ras le bol.

près de 700 détenus sont incarcérés à Fonds Sarail, alors que l’établissement a une capacité théorique d’accueil de 540 places. La surpopulation carcérale touche particulièrement le quartier de la maison d’arrêt pour hommes : actuellement, 126 prisonniers dorment sur des matelas posés à même le sol. Face à cette surpopulation, il y a un manque criant de moyens humains, notamment pour assurer la sécurité du site. Le cas de la Guadeloupe est loin d’être isolé, puisque la surpopulation carcérale est de plus de 200 % à Mayotte et de plus de 150 % en Guyane. Madame la ministre, le point d’alerte est atteint dans les centres pénitentiaires outre mer. Il est urgent d’agir. Que compte faire le Gouvernement face à cette situation, qui ne peut plus durer ? La parole

chaque jour par les surveillants pénitentiaires, parfois au péril de leur propre sécurité. L’agression, le 27 octobre dernier, d’un agent du centre pénitentiaire de Baie Mahault est un acte grave et inadmissible. La personne détenue responsable de cet incident a depuis lors été transférée vers un autre établissement pénitentiaire du territoire métropolitain. La direction des services pénitentiaires de l’outre mer a également pris des engagements auprès de l’intersyndicale, afin de trouver une réponse aux attentes des agents. À ce jour, 730 personnes sont incarcérées au centre pénitentiaire de Baie Mahault, pour un nombre de lits disponibles s’élevant à 620. Sur cette base, le taux de surpopulation carcérale global est de 149 %. La capacité théorique de l’établissement est en revanche de 490 cellules. Si le taux d’occupation du quartier centre de détention est optimal, le quartier maison d’arrêt souffre effectivement d’un taux très élevé, soit 196 %. La direction de l’administration pénitentiaire s’emploie depuis plusieurs années déjà à optimiser l’occupation des places disponibles dans les établissements et quartiers pour peine, afin de désengorger autant que possible les maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt. Cette stratégie, qui vise aussi des personnes détenues aux faibles reliquats de peine, porte ses fruits : le taux d’occupation de ces structures est passé de 87,3 % en 2020 à 98,5 % aujourd’hui, soit une hausse de plus de onze points en quatre Des transferts réguliers de personnes incarcérées depuis les établissements pénitentiaires ultramarins vers ceux de l’Hexagone continuent également. En termes de moyens humains, le centre pénitentiaire de Baie Mahault est dans une situation favorable, avec un taux de couverture des emplois du personnel de surveillance de 94 Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’Incarville, le garde des sceaux a également souhaité prioriser le renforcement de la présence d’équipes locales de sécurité pénitentiaire en outre mer. Quatre postes supplémentaires seront ainsi ouverts pour le centre pénitentiaire de Baie Mahault. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon l’ONU, la situation à Gaza est apocalyptique et des milliers de Palestiniens courent le risque imminent de mourir. Le système de santé est confronté à un effondrement total. Les structures de santé ont été en grande partie bombardées. Le personnel médical est une cible. Au mois de mai 2024, l’intensification des bombardements à Rafah et les ordres d’évacuation militaire ont entraîné, une nouvelle fois, le déplacement d’environ un un million de personnes. Selon l’Unicef, les familles déplacées vivent dans un dénuement total. Les conditions de vie sont indescriptibles : absence d’eau, de nourriture, de médicaments et de soins.

Où en sommes nous à ce jour ? Le 19 novembre 2023, le Président de la République avait annoncé qu’un porte hélicoptères configuré pour du soutien hospitalier, avec une capacité de quarante aurait vocation à traiter les cas les plus graves et à permettre la prise en compte de civils blessés, afin de les faire soigner dans les hôpitaux alentour si nécessaire. de l’occupation actuelle de ces quarante lits ?

M. le ministre délégué. Madame la sénatrice Poncet Monge, je vous remercie d’avoir rappelé l’engagement de la France et du Président de la République. Vous connaissez notre position constante

le, stationné en Égypte du 27 novembre 2023 au 27 janvier 2024, a permis la prise en charge de plus de 120 blessés dans un état grave. Le dispositif sanitaire a été mis en place en partenariat avec les autorités égyptiennes, les Nations unies, le Croissant Rouge égyptien, et avec le soutien de nombreux partenaires, notamment de l’Union européenne.

le soutien aux forces armées libanaises. Madame la sénatrice, notre engagement est collectif. Il est celui d’un pays qui sait combien sa sécurité est liée à celle du Proche Orient et qui est décidé à y faire entendre sa voix

Face à la hausse des implantations illégales dans des zones agricoles et inondables, la commune de Caumont sur Durance a établi un partenariat avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) visant à exercer un droit de préemption sur les terrains agricoles destinés à la vente qui ne sont pas acquis par des exploitants agricoles. agricoles. Cependant, des pratiques récentes ont mis en évidence des lacunes dans l’application de ce droit, notamment au travers de manœuvres visant à limiter son efficacité. En effet, des propriétaires cherchant à esquiver la préemption de leur terrain par les municipalités concluent des baux emphytéotiques. telle pratique soit légale, elle sert en l’espèce à perpétuer l’utilisation non conforme des terres agricoles. Face à un tel détournement du cadre légal, qui compromet tant les objectifs de protection des espaces agricoles que le respect de la régulation, comment

auprès de nos agriculteurs et viticulteurs, comme elle s’y était d’ailleurs engagée. Vous soulevez une question épineuse sur le caractère frauduleux des baux emphytéotiques. Il est en effet difficile de qualifier le caractère frauduleux d’un tel bail dans la perspective d’une préemption. La jurisprudence est venue apporter des précisions casuistiques. Elle indique notamment que, si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété en fin de contrat, ce dernier sera soumis au droit de préemption. Il appartient donc au notaire chargé d’établir le bail de déterminer si celui ci est soumis au droit de préemption. À cet égard, je ne puis que recommander à l’ensemble de la profession notariale la plus grande vigilance. Safer exercent leur droit de préemption conformément à leur mission, qui est de garantir le maintien de l’usage agricole. Le cahier des charges qu’elles demandent aux candidats repreneurs et l’étude qu’elles réalisent selon les priorités des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles contribuent également à cet objectif. Par ailleurs, les collectivités qui possèdent des pouvoirs d’aliénation peuvent les exercer sur des baux emphytéotiques ou se prémunir contre des constructions illicites en zone naturelle ou agricole. Il convient de souligner que ce pouvoir a été renforcé par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et

Comme vous le savez, une manifestation de grande ampleur a eu lieu au début de l’année 2024. Le gouvernement précédent s’était engagé à faire droit aux demandes légitimes de cette profession.

de la taxe foncière sur le non bâti. Le dispositif a prouvé son utilité. La procédure illustre la simplification attendue : aucune démarche du propriétaire ou de l’exploitant Par ailleurs, les demandes d’aide à la conversion en agriculture biologique pour la coriandre ont connu une hausse importante en 2024, particulièrement en Occitanie. Cette hausse est essentiellement liée au montant important de la prime associée à cette culture, sans lien avec une hausse de la demande de coriandre bio. Si la préfecture de région a appliqué un plafonnement à trois hectares sur les surfaces cultivées en coriandre, une exception a été apportée, afin de prendre en compte la situation des jeunes agriculteurs, pour lesquels le plafonnement a été rehaussé à neuf hectares.

Les aléas significatifs sont pris en charge par l’assurance récolte pour les exploitants ayant fait le choix de s’assurer. L’indemnisation se déclenche alors au delà de 20 % de pertes. Les primes d’assurance sont l’objet d’une subvention publique à hauteur de 70 %. Enfin, les aléas catastrophiques sont pris en charge par l’État, la solidarité nationale, pour tous les agriculteurs, assurés ou non. La parole

amplifiés par le changement climatique et par le recul de l’usage de produits phytosanitaires. Depuis quelques années, la filière viticole fait face, en Gironde et dans toute la France, à des aléas tels que le gel, la grêle ou les maladies cryptogamiques comme le mildiou, l’oïdium ou encore le black rot. Ces maladies, qui sont aggravées par l’humidité et par les vagues de chaleur, s’installent désormais régulièrement dans nos vignes, rendant le travail de nos viticulteurs toujours plus difficile. Aujourd’hui, il devient quasiment impossible de distinguer les dégâts liés au climat de ceux causés par les infections sanitaires. Aussi, les viticulteurs qui prennent la précaution de souscrire à une assurance climatique avec complémentaire sanitaire sont, de manière incompréhensible, pénalisés à double titre. D’un côté, un abattement sanitaire est systématiquement appliqué par l’État et les assureurs sur les indemnisations climatiques ; de l’autre, leur couverture sanitaire n’ouvre droit ni à la subvention de la politique agricole commune (PAC) ni au fonds de solidarité nationale (FSN). Monsieur le ministre, pourquoi cette injustice persistante ? Pourquoi la France ne reconnaît elle pas la nécessité d’inclure l’aléa sanitaire dans les conditions de soutien de la PAC et du fonds de solidarité nationale, alors même que l’Union européenne l’autorise

%. Si, pour les viticulteurs et agriculteurs qui souscrivent une double assurance climatique et sanitaire, les règles européennes excluent la possibilité d’ouvrir une expérimentation dérogatoire au plan stratégique national (PSN) de la France pour la PAC, pour la PAC, le Gouvernement est pleinement mobilisé face à la multiplication des aléas. La réforme de l’assurance récolte, mise en œuvre depuis 2023, a permis d’améliorer la prise en charge des aléas affectant les viticulteurs, qui peuvent tous bénéficier, désormais, de l’indemnisation de solidarité nationale.

Par ailleurs, l’État accompagne les viticulteurs dans leur effort de réduction de l’usage des produits phytosanitaires en travaillant au développement de solutions permettant de protéger les cultures dans ce contexte d’adaptation.

de nouvelles formes de contractualisation couvrant la prise de risque liée au changement des pratiques. La parole

Les autorisations de mise sur le marché ont donc été retirées et l’utilisation des stocks n’est plus permise. Aucune solution de substitution n’a cependant été trouvée pour permettre aux producteurs de maintenir leur activité, si ce n’est un désherbage manuel, extrêmement coûteux en main d’œuvre. La filière de la chicorée et la filière endivière font partie intégrante du patrimoine des Hauts de France, en particulier du département du Nord. La maîtrise des cultures est assurée par une filière structurée et implantée majoritairement dans les plaines de Flandre. Les étapes de la transformation de la plante sont assurées par plus de 200 planteurs, sécheurs et torréfacteurs, au moyen d’une technologie spécialisée et performante, qui garantit des produits sains et de qualité. Ces filières assurent à elles seules la quasi totalité de la production nationale et près d’un quart de la production mondiale. Elles sont donc source d’exportations pour la France. Pourtant, leur avenir est très incertain. incertain. Les professionnels sont bien conscients qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’autoriser le Bonalan, eu égard à son impact négatif pour notre planète ; ils ne le demandent d’ailleurs plus vraiment. Toutefois, monsieur le ministre, nous partageons tous le même mantra : « Pas d’interdiction sans solution !

de sécurité des aliments (AESA), qui a conclu, en 2019, que la substance ne répondait pas aux critères d’approbation de la réglementation actuelle. La France a alors mandaté l’AESA pour évaluer l’effet de diverses méthodes d’atténuation des risques, qui permettraient de maintenir l’approbation. a toutefois maintenu ses conclusions, ce qui a conduit la Commission européenne à ne pas renouveler l’approbation de la benfluraline. À la demande de la France, le délai de grâce maximal pour la distribution et l’utilisation des stocks de produits a été porté à quinze mois.

La filière a été tenue régulièrement informée de l’avancée des travaux européens et des initiatives prises par la France pour conserver un usage sûr. Afin d’anticiper la préparation au retrait de la benfluraline, une dérogation a été octroyée en avril 2024 pour expérimenter l’efficacité et la sélectivité En parallèle, une convention spécifique à hauteur de 100 000 euros a été signée avec l’Association des producteurs d’endives de France (Apef) pour la réalisation en 2024 et 2025 d’essais de désherbage avec des molécules de substitution. Les résultats obtenus avec plusieurs produits montrent que la benfluraline est substituable dans des conditions techniques acceptables. En 2025, il pourra être envisagé de reconduire les dérogations octroyées en 2024. Pour les perspectives moins immédiates, le désherbage des chicorées a été recensé parmi les usages prioritaires du plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes. L’Apef a en outre déposé une lettre d’intention pour conduire un projet dans le cadre du Parsada (plan d’action

Il était temps, car la colère de nos agriculteurs ne cesse, à juste titre, de monter ! J’apprends par ailleurs ce matin que de grandes surfaces vendent le litre de vin de côtes du rhône de qualité à 1,90 euro, alors que son coût de production est au moins 50 % plus Comment voulez vous que les viticulteurs s’y retrouvent ? Qu’en est il du dispositif d’arrachage viticole dans le Sud Est, ouvert le 15 octobre dernier ? Quand aura lieu sa mise en place concrète ? outre, n’est il pas conditionné à des usages de diversification destinés à la production alimentaire humaine ? Les remontées de terrain révèlent déjà que les structures viticoles les plus en difficulté risquent de devoir arracher la totalité de leurs vignes

Pour accompagner les agriculteurs face à ces défis, l’État finance des plans d’investissement visant à adapter l’agriculture au changement climatique dans le cadre de France 2030 et de la planification écologique. Il a également mis en place la réforme de l’assurance récolte pour accompagner économiquement les agriculteurs victimes de catastrophes climatiques.

En ce qui concerne les filières que vous citez, 3,6 millions d’euros ont bénéficié aux producteurs de cerises au titre de l’aide exceptionnelle mise en place en 2023. La filière a également bénéficié d’un guichet dédié permettant de financer des agroéquipements spécifiques pour accompagner la lutte contre les ravageurs et les conséquences du changement climatique.

Nous pouvons nous en féliciter, car cette coconstruction entre l’État et la filière a permis de définir, en complément de mesures d’urgence, des actions structurelles dont la filière avait besoin.

Et pendant que les constructeurs voient leurs commandes s’évaporer – la faute à des taux d’intérêt qui jouent les trouble fête –, nos concitoyens se voient exclus de la fête de l’accession à la propriété. C’est comme dans un bal où seuls les plus riches sont invités, tandis que les autres regardent par la fenêtre, l’air désemparé. Et que dire de cette obligation légale de trouver un assureur ? Avec la fragilité des constructeurs, ces garants jugent le risque trop élevé et ferment la porte au nez des chantiers. Résultat, les nouvelles constructions restent bloquées comme un vieux moteur qu’on ne pourrait redémarrer.

Je réclame le droit de rêver en construisant une jolie maison dans notre bourgade, le droit de m’émouvoir de son charme scintillant sans craindre une dérobade ! » Madame la ministre, il est grand temps de redonner le droit de rêver aux Français, et cela commence par débloquer la situation. Que comptez vous faire pour y parvenir ? La parole

Jean Michel Arnaud, et des logements classés E, dès 2034. Ces obligations s’appliqueront également – nous le savons depuis peu – aux meublés de tourisme. Sans remettre en cause la nécessité d’une décarbonation de nos politiques publiques, ce DPE pose plusieurs difficultés. Tout d’abord, les délais prévus se révèlent bien trop restreints au vu du temps de travaux nécessaire pour la mise en conformité des logements concernés. Ensuite, les calculs ne sont pas fiables, compte tenu de la diversité des situations, sans parler de la formation – hélas ! souvent défaillante – de certains professionnels.

j’ai constaté que, depuis quelques années, des entreprises proposaient des services de sous location et de conciergerie aux propriétaires de biens immobiliers. En contrepartie d’un loyer mensuel assuré et stable, ces entreprises réalisent des prestations de sous location de courte ou moyenne durée. Souvent proposées des plateformes en ligne, ces offres s’adressent en majorité à une clientèle touristique. Alors que la France pâtit d’un manque drastique de logements, ce nouveau procédé de sous location ne fait qu’accentuer le déséquilibre entre l’offre et la demande. Il a également des impacts fiscaux non négligeables.

substantielle. En outre, les communes appartenant au périmètre géographique de la taxe sur les logements vacants peuvent moduler de +5 % à +60 % la cotisation de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

les propriétaires de logements vacants, d’entrer en contact avec eux et de les informer sur les incitations à la remise sur le marché. Cet outil est utilisé à Paris depuis mars 2023, et nous ne pouvons que le saluer.

le prix des carburants en Guyane participe à la cherté de la vie et mobilise régulièrement élus et population en raison des niveaux records atteints. Par exemple, le sans plomb est actuellement vendu à 1,90 euro par litre, quand il coûte 1,72 euro dans l’Hexagone. l’Hexagone. Plus grave, nos voisins immédiats du Suriname, du Guyana et du Brésil le payent entre 94 centimes et 1,10 euro – moitié moins cher ! Ce constat posé, il faut réagir, et des solutions existent. Selon le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) de 2022, le marché des carburants aux Antilles et en Guyane est non pas un système de prix administrés, mais un triple monopole au bénéfice d’une entreprise, la Sara monopole sur l’importation des produits pétroliers, ainsi que sur le raffinage et le stockage. Selon ce même rapport, l’arrêt de l’activité de raffinage serait la seule solution pour permettre une baisse significative des prix, de l’ordre de 14 centimes d’euro à 18 centimes d’euro. Monsieur le ministre, qu’en est il de cette proposition et de toutes les autres qui sont contenues dans ce rapport ? Quelle est la légitimité d’un système dans lequel l’État garantit 23 millions d’euros de rémunération à l’actionnaire de la Sara, tout en acceptant des prix élevés pour le consommateur ? Enfin, ce gain de 14 centimes à 18 centimes laisserait la Guyane encore loin des prix pratiqués par ses voisins, en particulier sur le plateau des Guyanes. Tous sont producteurs de pétrole. N’y a t il pas là une double peine pour la Guyane ? Elle ne peut importer à moindre coût les carburants de ses voisins et doit le faire depuis l’Europe. Il lui est également interdit d’exploiter le pétrole présent dans son sous sol au titre de la loi Hulot, alors même que ce texte n’a pas interdit de nouveaux forages en Gironde en 2023 et que l’Europe achète la moitié de la production pétrolière du Guyana… Monsieur le ministre, n’est il pas temps de mettre fin à cette hypocrisie et d’abroger la loi Hulot pour la Guyane ?

Si ces prix réglementés sont aujourd’hui proches de ceux qui sont constatés dans l’Hexagone, des marges de progrès importantes ont été mises en exergue, à la fois aux Antilles et en Guyane. L’IGF a ainsi établi des pistes de travail destinées à favoriser une meilleure transparence dans la définition de ces prix. C’est ce que je souhaite également faire sur la question de la vie chère – nous en avons déjà parlé ensemble il y a quelques semaines. Elle a également préconisé de réexaminer plusieurs éléments de calcul des prix des carburants, du fonctionnement et donc de la de la rémunération de la Sara. C’est pourquoi une réforme de la régulation des prix et du système de distribution a été actée au moment du comité

Un fonctionnaire absent, c’est la double peine pour les Français. D’un côté, on recrute de nouveaux fonctionnaires : je rappelle que plus d’un million d’agents ont été recrutés entre l’an 2000 et aujourd’hui. Et pour quels résultats, alors que 51 % des Français disent ne pas être satisfaits de leurs services publics, selon une étude de l’Ifop,

ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont en cause, mais les gestionnaires. Paris en est le symbole ! La Ville de Paris emploie plus de personnes que toutes les institutions européennes

que je recevrai dès jeudi après midi : de meilleures conditions de travail – cela peut évidemment avoir un impact sur l’absentéisme ; moins de bureaucratie pour les agents, en essayant de leur faciliter la tâche, pour qu’ils puissent chaque matin être heureux d’aller au travail et se concentrer sur leur cœur de métier ; enfin, une meilleure protection fonctionnelle,